La séance est reprise. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à démocratiser le sport en France.

c'est ainsi que la démocratisation du sport en France pourra grandir. C'est un critère qui nous semble indispensable pour le classement Elo. Il y a un enjeu majeur à garantir, notamment, l'accès de l'audiovisuel public à ces événements, afin de ne pas confier cette diffusion à un marché trop restreint,

soient librement mis à disposition du public, à la condition que cette mise à disposition ne fasse l'objet d'aucune contrepartie financière. Nous connaissons tous des sites internet

comme le fait la loi de 2000, protéger les collectivités. Je ne comprends pas que vous, représentants des collectivités, puissiez être contre, compte tenu des dérives observées dans le financement de certains clubs professionnels par certaines collectivités.

2016, outre les interdictions administratives et judiciaires de stade, le législateur a doté les clubs et organisateurs d'événements sportifs d'un pouvoir d'interdiction commerciale de stade. Autrement dit, on a une nouvelle fois externalisé un pouvoir de sanction, sans en définir strictement les contours. Ainsi, et en théorie, au seul motif qu'il cherche à préserver sa sécurité, un club peut refuser de vendre un billet à un supporter

Une telle procédure amiable est d'autant plus nécessaire pour les clubs qu'ils s'exposent, en l'occurrence, à une condamnation ultérieure

du maintien de l'ordre. Il convient donc de mieux borner les ICS, en les limitant dans le temps et en les formalisant davantage. : La parole est à M. Stéphane Piednoir. Comme vous le savez, les juges et les préfets peuvent interdire de stade un supporter coupable d'un comportement portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Les organisateurs de manifestations sportives peuvent soit déposer plainte et se constituer partie civile devant un tribunal, soit écrire au préfet pour signaler le comportement de ce supporter. si ni le procureur ni le préfet considère qu'il faut y donner suite, il serait incompréhensible qu'une société commerciale puisse se substituer à l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire et à l'appréciation régalienne de l'autorité de police.

parole est à M. Thomas Dossus. Les ICS, qui ont été créées en 2016, permettent aux clubs de refuser l'accès au stade aux personnes qui contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité. Nous ne sommes pas opposés par principe aux ICS, mais nous souhaitons,

En 2007, le Conseil d'État a rendu un avis indiquant que les clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, ont une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité lors du déroulement des rencontres.

imposée aux clubs par une obligation de moyens.

viennent de défendre. Dans les faits, l'obligation de résultat imposée aux clubs est intenable. C'est pourquoi le présent amendement tend à lui substituer une obligation de moyens, qui permettrait à la commission de discipline de retrouver une marge d'appréciation et de sanction graduée entre les clubs irréprochables et les clubs plus négligents.

Mme Sabine Van Heghe. Cet amendement tend à limiter les motifs d'interdiction administrative de stade, dès lors qu'une personne constitue une menace grave pour l'ordre public.

: La parole est à Mme Marie Mercier. Les interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées dans 75 % des cas, du fait notamment d'erreurs dans l'identification du supporter auteur du comportement reproché.

je comprends l'intérêt de mieux circonscrire les interdictions administratives de stade, mais on ne saurait envisager de réduire les outils pour lutter contre les violences dans les stades. L'avis de

ce qui démontre que leur usage est encore à parfaire. Il est donc indispensable que le juge administratif puisse se prononcer rapidement sur des arrêtés emportant des conséquences aussi lourdes en matière de libertés individuelles, de respect de la vie familiale et d'activité professionnelle.

l'heure actuelle, il est inscrit dans la loi qu'un recours pour excès de pouvoir contre une sanction administrative peut être assorti d'un recours en référé, lorsque certaines conditions sont satisfaites- lorsque l'urgence le justifie, ou bien qu'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il est donc tout à fait possible pour les supporters qui seraient soumis à une interdiction administrative illégale de bénéficier d'un recours rapide en vue de la suspension de la mesure. Cela dit, mesdames, messieurs

restons dans le même esprit, évoquant la problématique de la proportionnalité et des libertés individuelles. L'interdiction administrative de stade est prise par simple arrêté préfectoral. La personne visée n'a pas la possibilité de se défendre. la saisie du juge administratif est quasi systématique, comme on le constate aujourd'hui. Nous proposons que le juge puisse se prononcer très rapidement, afin d'éviter ces mesures privatives de liberté sur des durées excessivement longues, qui représentent, je l'ai dit à l'instant, jusqu'à 50 ou 60 obligations de pointage au commissariat par an.

Si nous proposons de fixer une échéance à trois semaines avant les déplacements prévus, nous proposons aussi que le préfet puisse, par dérogation, se soustraire à cette obligation. En effet, on peut entendre qu'une situation d'urgence ou un événement du week-end précédent justifie une mesure dérogatoire, mais il nous semble essentiel de fixer un cadre. Ainsi, en 2014, les supporters lensois ont été interdits de déplacement à Bastia, le préfet invoquant des événements ayant eu lieu

Ce sujet des déplacements collectifs devient de plus en plus central, ne serait-ce que parce que leur nombre a connu une hausse de 6 700 en quatre ans ! Cette augmentation est due, à la fois, à l'état d'urgence consécutif aux attentats de Paris et à l'application d'interdictions au niveau amateur. Il est tout de même plus simple d'encadrer

La mise en place de dialogues préalables pourrait permettre de mieux encadrer et organiser les déplacements, tout en responsabilisant à la fois les pouvoirs publics, les clubs et les groupes de supporters. L'amendement

d'interdire le déplacement de supporters de clubs visiteurs dans la commune ou aux abords du stade du club recevant la manifestation sportive. Il donne lieu, aujourd'hui, à un usage croissant et pas toujours justifié-

Enfin, nous souhaitons que la Division nationale de lutte contre le hooliganisme soit associée à ces discussions, afin que l'expertise de cette institution reconnue puisse être prise en compte. L'amendement n° 46 rectifié,

hélas, qu'il faut moins de membres des forces de l'ordre pour encadrer un déplacement organisé que pour faire appliquer un arrêté d'interdiction de déplacement. Il est parfois plus aisé

Mandelli. Le présent amendement a pour objet d'encadrer le mécanisme permettant au ministre de l'intérieur, au représentant de l'État ou au préfet de police d'interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporters d'une équipe sur les lieux d'une manifestation sportive. Sauf circonstances exceptionnelles, il est proposé que l'arrêté intervienne au moins trois semaines avant la manifestation.

voulue et souhaitée par les associations de supporters, se traduit par cette décision, prise en concertation avec le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux. Il s'agit de punir ceux qui tentent d'introduire des objets potentiellement dangereux dans les stades. C'est un moyen dissuasif,

messieurs les sénateurs, appelons de nos voeux. Il faut commencer par assumer nos responsabilités, en garantissant au préalable la sûreté de nos enceintes sportives pour tous les spectateurs

En effet, les décisions jurisprudentielles pour la détention et l'usage de fumigènes ou de fusées oscillent aujourd'hui entre le rappel à la loi et des amendes avec sursis aux montants trois à quatre fois inférieurs à 800 euros. L'augmentation proposée du montant de l'amende forfaitaire, qui serait fixée

important d'aller plus loin en autorisant complètement l'usage des fumigènes, et cela pour plusieurs raisons. Comme le rappelle le rapport de Marie-George Buffet et de Sacha Houlié, le caractère dangereux des fumigènes résulte aujourd'hui de leur interdiction, qui conduit les supporters à les allumer en se dissimulant notamment sous des bâches qui ne sont pas ignifugées. De la même manière, alors que la détention ou l'usage

et la répression mises en oeuvre depuis des années ne servent à rien, l'usage des fumigènes n'ayant jamais été aussi répandu. D'ailleurs, je note une une certaine hypocrisie sur le sujet, puisque, si vous regardez la plupart des images et des clips de promotion des compétitions professionnelles, celles-ci intègrent systématiquement une tribune où des fumigènes soulignent l'ambiance du stade. Il est regrettable qu'en matière de fumigènes les pouvoirs publics soient pour le coup à contretemps des supporters, mais aussi des clubs, dont la plupart ont indiqué qu'ils les acceptaient tant qu'ils pas détournés de leur usage normal, créant des dommages aux biens et aux personnes qui engagent la responsabilité du supporter. D'ailleurs, de nombreux clubs ont déjà fait le choix de négocier, dans le cadre de l'expérimentation des fumigènes, avec les supporters

commission ? La nouvelle rédaction de l'article 11 A ouvre la voie à un usage autorisé des fumigènes. C'est une avancée suffisante, dont il conviendra d'évaluer les résultats. Il ne m'apparaît pas opportun d'aller au-delà en autorisant sans condition leur usage dans les stades. La commission émet donc un avis défavorable.

feux rouges ; moi, je vous parle de fumigènes ! Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Vous savez comme moi que les sanctions sont complètement disproportionnées,

Paralympiques de 2024. Une compétition doit être organisée en marge des JO. Cet amendement vise à contrôler l'honorabilité des encadrants professionnels et bénévoles d'activités e-sportives, notamment les encadrants de mineurs, sur le même modèle que ce qui existe pour les activités sportives. L'essor du e-sport en France doit être encadré,, sur les questions d'honorabilité. En effet, le risque existe que des encadrants sportifs interdits d'exercice, car ils sont dangereux notamment pour les mineurs, puissent se reconvertir dans le e-sport. C'est pourquoi il est nécessaire de donner les moyens aux structures d'accueil de réaliser les mêmes contrôles que dans le milieu sportif. Cela permettra notamment de sécuriser le développement du e-sport, et de le soutenir. Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application du présent article, pour sécuriser les acteurs et mettre en place les modalités de mise en oeuvre du contrôle. Quel est l'avis de la commission

qui sont principalement les sports collectifs, ou dans d'autres sports, puisque les exigences de performance vis-à-vis de ces derniers n'ont pas à être hiérarchisées. Elles pourraient même être interprétées par les arbitres des sports non professionnels comme de la condescendance. Ensuite, le parcours d'accès à l'excellence sportive dans les activités arbitrales, qui relève du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, prend déjà en compte, dans chaque discipline, les enjeux de formation initiale et de reconversion professionnelle de cette population. Les fédérations sont ainsi bien sûr compétentes pour déterminer leur stratégie d'inscription des arbitres, y compris ceux qui officient dans les divisions professionnelles sur les listes de haut niveau. Enfin, il nous semble dangereux de prévoir dans la loi la conclusion obligatoire d'une convention entre la fédération et l'arbitre de sport professionnel,

relatives à la liste des juges et arbitres de haut niveau, quelles que soient les divisions dans lesquelles ils officient. Je précise que l'amendement adopté en commission ne résulte pas d'une demande de l'Association française du corps arbitral multisports (Afcam).

le présent article. Il vise à donner un statut aux juges et aux arbitres de haut niveau, qui sont aujourd'hui identifiés par la liste dont parlait à l'instant Mme la ministre.

En outre, vous confondez les divisions professionnelles dans lesquelles évoluent ces arbitres et les arbitres qui exercent cette activité à titre professionnel exclusif.

les sols sportifs et les aires de jeux ou de loisirs. Ces entreprises sont fortement impliquées dans la promotion et la valorisation des infrastructures et des lieux de pratiques sportives et de loisirs, en particulier auprès des collectivités territoriales.

Le tissu économique local participe en effet au soutien financier à la mobilité des jeunes sportifs ultramarins. D'ailleurs, en 2018, le ministère des outre-mer soulignait la participation d'entreprises ultramarines à ce financement, l'alimentation du fonds d'expérimentation pour la jeunesse (FEJ) par des entreprises en zone franche d'activité. Les mécanismes de déductibilité fiscale sont également une incitation aux efforts financiers du secteur privé.

constatation des faits, et non de leur réalisation, ce qui laisse un temps suffisant à l'administration pour faire usage d'une telle mesure. Les mesures de police administrative sont des dispositions d'urgence, prises en attendant que l'autorité judiciaire engage une procédure et prononce une interdiction de stade. Elles ne peuvent pas s'entendre comme des sanctions prises plus de deux mois après la constatation des faits.

le dernier d'une longue série ! Par sa circulaire du 18 novembre 2019, le ministre de l'intérieur demandait aux préfets de se fonder sur la particulière gravité des antécédents pour justifier de la nécessité

dans le cadre d'un parcours médical, ou encore au développement de la pratique libre, que l'on va encourager en ouvrant largement les infrastructures. Je salue

soutenu le développement du sport en entreprise, en imposant la création de douches dans les nouveaux locaux et en inscrivant le sport dans les matières négociées chaque année entre les salariés et les employeurs. la réaffirmation ferme des objectifs de lutte contre toutes les formes de violence dans le sport, à la création d'une charte nationale du bénévolat sportif, à l'interdiction des certificats de complaisance et du port de signes religieux ostensibles dans les compétitions sportives, à la rationalisation des règles de nouvelle gouvernance, la création d'un débat entre les fédérations sur la rémunération des présidents, au renforcement des contrôles éthiques, au soutien au sport professionnel l'encadrement des sociétés commerciales,

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.